La séance est ouverte.

et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, gaz, électricité, carburants : depuis plusieurs mois, les Français font face à des hausses importantes des prix qui mettent en difficulté les plus modestes à l'approche de l'hiver. Ces augmentations s'ajoutent aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui ont touché en premier lieu les plus fragiles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de l'année, le montant mensuel du tarif réglementé du gaz a augmenté de 50,8 les tarifs réglementés de l'électricité devraient bondir de 12 % en début d'année et le prix du sans plomb 95 a retrouvé son niveau d'octobre 2018, juste avant la crise des « gilets jaunes Certes, des éléments conjoncturels liés à la reprise économique mondiale expliquent ces tensions sur les prix, avec une demande en forte hausse. Les facteurs de formation des prix, avec le poids des taxes, accentuent également l'élasticité des tarifs. La situation illustre aussi la difficulté de l'Union européenne à mettre en place, dans le contexte de la transition écologique, une stratégie énergétique commune profitable aux citoyens européens, alors que les intérêts des États membres sont souvent divergents. Néanmoins, par-delà ces questions, l'urgence demeure pour nos concitoyens. Vous avez annoncé la mise en place d'un « bouclier tarifaire » pour contenir, d'ici au printemps 2022, la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Vous envisagez également de relever au besoin le chèque énergie. Si ces décisions sont un premier pas que nous saluons, elles restent ponctuelles. Elles ne suffiront pas en cas d'hiver rigoureux ou de nouveau choc d'offre ou de demande. Plus largement, c'est bien notre souveraineté énergétique qui est en jeu, la seule à même, grâce à notre mix, de garantir que l'énergie reste un bien commun accessible. Comment comptez-vous donc agir pour que l'énergie ne devienne pas, à long terme, un facteur d'inégalités qui grèverait le pouvoir d'achat des Français ? La parole

hausse du fait de l'augmentation du prix du gaz liée à l'accroissement de la demande suscitée par la reprise mondiale ainsi qu'à une réduction de certaines productions, notamment en Russie et en Norvège. Face à cette situation largement due à des facteurs extérieurs, il nous fallait effectivement des réponses pour les ménages. Ainsi, une aide sociale supplémentaire de 100 euros en faveur des quelque nous allons déployer ce bouclier tarifaire qui vise à protéger tous les Français. Les prix du gaz seront bloqués tout l'hiver à leur niveau d'octobre. Sans cela, la facture des Français aurait pu augmenter de 30 %. S'agissant de l'électricité, l'augmentation des tarifs réglementés sera au maximum de 4 % par rapport à 2021, soit environ 5 euros par mois

S'agissant du gaz, quand les prix baisseront- sans doute au printemps -, nous diminuerons un peu plus lentement les tarifs afin de revenir à la normale. Il s'agit d'un lissage, à la montée comme à la descente, de manière à en amoindrir les effets pour les ménages français.

le 30 septembre, sans attendre que le Conseil d'État ait rendu son jugement sur le fond, sortait le décret d'application de la réforme de l'assurance chômage. Le Conseil d'État avait pourtant suspendu la réforme, considérant que son application constituait « une erreur manifeste de jugement eu égard à la conjoncture économique. Vous répondez que les critères de retour à bonne fortune sont désormais remplis et permettent aux demandeurs d'emploi de privilégier les emplois stables et non les parcours d'emploi fractionnés qu'ils privilégiaient, selon vous, du fait d'une allocation trop généreuse. Sur vos deux critères de retour à bonne fortune, pouvez-vous alors nous indiquer quelle est la part d'embauches en contrats de plus de quatre mois, voire six mois, période désormais requise pour l'indemnisation ? Combien sont en CDI, alors que de multiples lois ont favorisé le recours aux contrats précaires ? S'agissant de la baisse des chômeurs de catégorie A, encore faudrait-il compléter ce critère avec l'évolution à la hausse des catégories B et C, où se trouvent les salariés qui seront les plus affectés par votre réforme, et de la catégorie D, où atterrissent les contrats de sécurisation professionnelle à la suite de licenciements économiques, comme beaucoup de jeunes du dispositif « 1 jeune, 1 solution » ? Madame la ministre, quelles sont la pertinence et la robustesse de vos critères de retour à bonne fortune, au regard de la seule justification de la réforme de favoriser l'emploi durable,

En particulier, un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage s'applique, mais uniquement aux demandeurs d'emploi inscrits depuis cette date. En effet, nous pensons que la situation économique et la situation du marché du travail justifient pleinement la mise en oeuvre de cette réforme de l'assurance chômage. Vous le savez, nous avons eu 2,4 millions d'embauches ces trois derniers mois, ce qui est un record historique depuis au moins quinze ans. Je rappelle, par ailleurs, qu'on a 320 000 demandeurs d'emploi de catégorie A de moins

aux contrats courts avec le système de bonus-malus qui doit conduire les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs. Par ailleurs, nous voulons aussi encourager ceux qui le peuvent à travailler davantage : c'est le sens du nouveau mode de calcul

Alors que se négocient au niveau européen les seuils d'émissions de CO2 de certaines activités économiques qui entreront dans cette classification, et donc bénéficieront de financements verts et d'aides européennes, notre questionnement, notamment quant aux investissements, s'intensifie à l'approche de la fin de l'année. Le nucléaire est une filière historique, mais, surtout, d'excellence française. Elle nous garantit une part de souveraineté énergétique dont toute l'Europe bénéficie, y compris ceux de nos voisins qui mettent leur mouchoir sur leur mauvaise conscience d'importateurs d'électricité nucléaire. Cette énergie a toute sa place dans notre mix énergétique, même si sa part doit diminuer. C'est pourquoi la mobilisation des capitaux nécessaires afin de réaliser des investissements qui le sont tout autant ne peut être entravée. Surtout lorsque les experts ne convergent pas pour démontrer que cette énergie serait préjudiciable à l'atteinte de nos objectifs environnementaux ou à notre combat ultralégitime contre les effets du dérèglement climatique. climatique. La neutralité carbone en 2050 ne pourra pas se faire sans cette technologie bas-carbone. Y consacrer des moyens suffisants revient à financer la recherche pour maintenir sur l'existant des unités toujours plus fiables et efficaces. Enfin, cela signifie surtout se mettre en capacité d'accroître la sûreté des sites et de mieux garantir leur longévité. Les enjeux économiques et industriels sont immenses pour notre pays. Je prends pour exemple la centrale de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Prolonger son activité dans les meilleures conditions assure de garder un haut niveau d'expertise, une verticalité nécessaire dans tous les métiers sur site et sécurise l'évolution de notre mix énergétique. Madame la ministre, le temps presse. Je sais le Gouvernement investi. Pouvez-vous nous donner l'état des discussions après l'Eurogroupe d'hier et les positions que la France défendra dans les prochains mois ? Très bonne

Madame la sénatrice Paoli-Gagin, merci de rappeler le caractère absolument stratégique de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique. Cette énergie est stratégique, car, vous l'avez très bien dit, c'est une énergie indispensable pour décarboner notre économie.

Le nucléaire doit figurer dans la taxonomie. C'est le propos que nous portons, Barbara Pompili, Bruno Le Maire, Clément Beaune et moi-même dans tous nos conseils : conseil compétitivité, conseil climat, et financières (Écofin). Bruno Le Maire l'a encore porté en début de semaine de manière très nette et très précise. Très bien ! C'est dans cette direction que nous allons poursuivre les négociations avec fermeté, avec fermeté, parce que les faits sont têtus : on ne luttera pas contre le réchauffement climatique sans énergie nucléaire, ce qui n'est évidemment pas contradictoire évidemment pas contradictoire avec le fait de développer massivement les énergies renouvelables. Notre stratégie est fondée sur deux piliers : les énergies nucléaires et les énergies renouvelables. La parole

Monsieur le Premier ministre, une mission d'information sénatoriale vient de commettre un rapport sur les influences étrangères extraeuropéennes au sein de nos universités et du monde académique français. Il en ressort que des pays étrangers qui ne sont pas démocratiques ou qui ne partagent pas nos valeurs- je veux parler de la Chine, de la Russie ou de la Turquie -se livrent aujourd'hui à de véritables ingérences dans notre monde académique. Ils affectent des moyens considérables au service de leurs influences. influences. Ressort également qu'en France, les moyens mis à disposition pour connaître, comprendre et lutter contre ces ingérences ne sont plus aujourd'hui totalement adaptés à l'importance du phénomène. comment, par exemple, surveiller un institut Confucius hébergé dans une université ? On sait désormais que ces instituts ne sont pas là uniquement pour enseigner le chinois ou valoriser la culture chinoise, mais qu'ils se livrent à de véritables exercices d'influence dans les universités qui les hébergent. Comment protéger une communauté scientifique qui travaille sur la présence des chrétiens en Orient, sur le génocide arménien de 1916, alors que l'accès par le gouvernement turc au territoire et aux archives turques n'est plus facilité ? Cette communauté scientifique subit même parfois des pressions et des menaces inadmissibles. Monsieur le Premier ministre, l'intégrité scientifique et les libertés académiques sont des marqueurs essentiels dans nos démocraties occidentales. Ce sont des marqueurs essentiels pour nos libertés. Le Gouvernement l'entend-il de la sorte et comment entend-il mieux les protéger ?

touche un sujet majeur. C'est un sujet qui touche en réalité notre société dans son ensemble, mais qui appelle un traitement particulier s'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les vingt-six propositions que vous avez faites, visant cinq grands objectifs, font déjà l'objet d'un travail d'analyse approfondi et rigoureux de la part de mes équipes. Je tiens à rappeler, comme j'ai pu le faire lors de mon audition au mois de septembre, qu'effectivement il nous faut absolument préserver l'intégrité scientifique et la liberté académique, qui sont indissociables. C'est tout l'objet du deuxième objectif de votre rapport et c'est aussi ce que vous avez souhaité faire dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, qui contient des avancées majeures en la matière. Cet attachement aux libertés académiques et à l'intégrité scientifique ne doit évidemment pas limiter les interactions et les échanges internationaux, mais ceux-ci doivent se réaliser sans naïveté. Grâce au haut fonctionnaire de défense et de sécurité, à la mission ministérielle sûreté et sécurisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux 160 fonctionnaires de sécurité défense, au réseau coordonné, au dispositif de protection du potentiel scientifique et technique- nous portons un intérêt tout particulier à la recommandation de la mission qui vise à l'étendre à l'ensemble des disciplines universitaires-, nous nous sommes sommes emparés de ce sujet. Les conclusions et recommandations de la mission d'information du Sénat convergent très largement avec l'action de mon ministère et, plus largement, celle de ce gouvernement, en lien avec l'ensemble des administrations concernées. Vous ne

du fait des actions d'influence menées par ces pays qui ne partagent pas nos valeurs démocratiques, des phénomènes considérables contre lesquels on ne peut pas lutter avec un sabre de bois. » Nous sommes donc à la disposition du Gouvernement pour échanger sur ce sujet particulièrement grave.

Tout va bien, dormons tranquilles, puisque, quarante-huit heures après ces révélations, l'Union européenne supprime trois territoires de la liste des territoires non coopératifs. Trois paradis fiscaux de moins, c'est vrai que c'est un mauvais. La France allant présider le Conseil européen, monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale alors que notre dette flambe ? Pendant que certains cachent des millions dans les paradis fiscaux, nos étudiants font la queue devant les banques alimentaires et nos agriculteurs se débattent dans des difficultés infernales ? La parole

600 journalistes, 117 pays concernés et 12 millions de données qui seraient exploités ou exploitables par ce consortium de journalistes pour mettre au jour des pratiques d'optimisation, d'évasion, voire de fraude fiscale dans un grand nombre de pays, par le biais de sociétés offshore.

diligenter les contrôles fiscaux les plus sévères qui soient et de mettre en oeuvre, en lien avec le ministère de la justice, les sanctions et procédures judiciaires qui s'avéreraient les plus utiles. Nous continuons à oeuvrer contre la fraude fiscale, à la fois à l'échelle française et à l'échelle européenne. Nous avons permis l'adoption d'une loi de lutte contre la fraude en octobre 2018- vous aviez été active dans ces débats, -avec la création d'une police fiscale. Nous avons renforcé notre système d'information avec, notamment, la pérennisation de la rémunération des aviseurs fiscaux. Enfin, nous développons au niveau européen, sens dans lequel nous poussons, des échanges d'informations extrêmement poussés. Ainsi, pour 2019, ce sont 107 milliards d'euros de revenus fiscaux complémentaires à l'échelle de l'Union européenne qui ont été trouvés et dégagés par des échanges d'informations portant sur plus de 84 millions de comptes que nous avons pu ainsi investiguer et vérifier. Il y aurait Il y aurait beaucoup à dire pour développer les différents sujets et priorités que nous avons. Je crois pouvoir revenir, à l'occasion de prochaines questions, sur ce que nous faisons aussi en matière de lutte contre la fraude fiscale, et je veux vous assurer de ma détermination la plus totale à lutter contre cette fraude et à exploiter l'ensemble des données auxquelles nous aurons accès par les révélations que vous avez citées. Mme Nathalie Goulet, pour la réplique. Monsieur le ministre, nous sommes toujours dans l'. Votre bilan n'est pas exactement celui que vous dites : vous avez réduit les moyens humains pour le contrôle fiscal et douanier, vous avez démantelé la délégation nationale à la lutte contre la fraude, vous avez perdu du temps pour la mise en place du système de détection précoce de fraude à la TVA- c'est un système de (TNA) appliqué par tous les pays européens dont on vous a demandé depuis plusieurs années l'application en France, et qui vient seulement de l'être. Je rappelle que la fraude à la TVA représente 5 milliards d'euros détectés l'année dernière et 10 milliards au niveau de l'Europe. Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement du Sénat qui visait à interdire les aides covid aux entreprises disposant de filiales dans les paradis fiscaux, préférant- allons savoir pourquoi -la circulaire, qui est peut-être mieux que la loi. Vous me le direz peut-être. Il reste 777 enquêtes préliminaires actuellement ouvertes pour des affaires de fraude fiscale et de blanchiment. Vous vous êtes opposé à la position légitime du Sénat, qui a voté la possibilité de prolongation de ces enquêtes pour ces faits. Délai que vous vouliez réduire sans distinguo dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Enfin, pour mener ces enquêtes préliminaires, on ne compte que trois enquêteurs. Je ne suis pas certaine que l'adéquation soit exacte. Les chiffres publiés attestent de ce bilan désastreux. Le résultat de la lutte contre la fraude a été divisé par deux en 2017.

l'existence de 55 000 sociétés offshore détenant 6 500 milliards d'euros d'actifs au Luxembourg. Cette semaine, un consortium de journalistes publie une nouvelle enquête, les- bien que la boîte de Pandore ait été ouverte il y a déjà bien longtemps -par laquelle nous apprenons que 29 000 autres sociétés offshore viennent d'être mises au jour, créées et gérées par quatorze cabinets et officines spécialisés. M. le ministre Bruno Le Maire s'est déclaré « choqué », quand tous nos concitoyens sont ulcérés par ces révélations incessantes faites par la presse ces dernières années. Pour les milliardaires concernés, responsables politiques de très haut niveau, sportifs et trafiquants en tout genre, l'objectif est d'échapper à l'impôt et aux juges grâce à cette industrie de l'opacité. Le problème est systémique. Monsieur le ministre, comptez-vous en rester au choc et à la vérification ?

Il faut rendre à César ce qui est à César : le développement des outils de lutte contre la fraude fiscale date de plusieurs années. Lorsque l'on regarde les quelques années écoulées, on peut citer la loi relative à la

sur celle dite des. En la matière, l'administration fiscale française a identifié un certain nombre de contribuables français concernés, nous avons mené à leur terme 657 dossiers soit de régularisation, soit de redressement, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une judiciarisation. Cela a permis à l'État français de recouvrer plus de 200 millions d'euros

L'essentiel, pour moi, c'est que l'administration est au travail et que, quand elle travaille, cela paie et permet de sanctionner les fraudeurs. pour la réplique. Ces scandales successifs qui se traduisent à chaque fois par des milliards en fuite pour la République nécessitent une réaction déterminée. Vous le savez, nous sommes constructifs et nous nous permettons de vous suggérer trois pistes d'action immédiate. Premièrement, vous pouvez recréer des postes de contrôleur dès le projet de loi de finances qui vient devant le Parlement dans quelques jours. Pour rappel, 38 000 emplois ont été supprimés depuis 2002 dans les finances publiques. vous pouvez créer l'observatoire de la lutte contre la fraude fiscale, annoncé en 2018, jamais mis en place. Nous sommes candidats à titre bénévole. Troisièmement, la France va présider le Conseil de l'Union européenne à partir de janvier 2022. L'Union européenne a décidé hier de retirer de la liste des paradis fiscaux les Seychelles, en plein coeur des révélations du dernier scandale. Inscrivez à l'agenda de ce semestre une mise à jour de cette liste en y incluant notamment le Luxembourg et Chypre.

Beaucoup l'ont reconnu et ont salué cet effort sans précédent, mais certains ont choisi, il y a quelques jours, d'alimenter la polémique, en dénonçant une baisse de 50 millions d'euros des dotations, ce qui témoignerait selon eux d'un mépris du Gouvernement à leur endroit. Cette polémique est censée nous faire oublier l'ensemble des efforts financiers consentis par l'État durant la crise, alors même que le sujet de la discorde représenterait au total moins de 0,2 % du budget des régions.

que nous avons pu lire avec un certain étonnement que les régions et le Gouvernement ne semblaient pas partager la même vision de la réalité du pays. On comprend mieux ce slogan quand on sait que, parmi les actuels présidents de région, pas moins de deux sont déjà candidats à l'élection présidentielle, mais on peut douter que de telles déclarations servent la clarté et la sincérité du débat public. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler l'ensemble des mesures prises durant la crise pour soutenir les finances des collectivités locales et, singulièrement, celles des régions dans l'Hexagone comme en outre-mer ? La parole

Pour les régions d'outre-mer, l'effort de l'État s'est traduit par l'intégration dans le panier des ressources garanties des recettes liées à l'octroi de mer et à la taxe spéciale de consommation sur les carburants, ce qui représente un montant supplémentaire de 80 millions d'euros.

Merci, monsieur le président. C'est un honneur de représenter les Françaises et les Français établis hors de France au sein de notre assemblée. Mes chers collègues, il y a un an jour pour jour, notre compatriote Emmanuelle Charpentier recevait le prix Nobel de chimie. Établie hors de France depuis vingt-quatre ans, elle déclarait alors : « Je pense que la France aurait du mal à me donner les moyens que j'ai en Allemagne. La recherche scientifique a besoin d'être soutenue par le Gouvernement. » Un an plus tard, le constat est sans appel. La semaine dernière, le journal publiait une enquête accablante sur le déclin de la recherche en France, qui mettait en relief des moyens en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, des salaires indignes, des équipements vieillissants, ainsi que la dégradation des conditions de travail qui affecte la productivité de la recherche française. Loin de régler le problème, la loi de programmation de la recherche (LPR) votée en 2020 consacre le manque d'ambition du Gouvernement, en accroissant la précarisation des contrats et les inégalités entre laboratoires. En tant que conseiller consulaire et désormais sénateur représentant les Français de l'étranger, j'ai rencontré des centaines de compatriotes, doctorantes et doctorants, chercheuses et chercheurs, qui, devant ce manque cruel de moyens, ont fait le choix d'exercer leur métier et de vivre leur passion à Washington, à Cambridge, à Belém ou encore à Sydney. À l'heure ou la planète est confrontée à des bouleversements climatiques et sanitaires majeurs, comment le Gouvernement compte-t-il donner à la recherche française les moyens de répondre à l'urgence ? La parole

Madame la ministre, je constate que votre réponse n'est vraiment pas à la hauteur de l'urgence des défis climatiques et sanitaires auxquels nous devons faire face. Concernant le budget 2022, les augmentations annoncées sont très en deçà de ce qui était prévu dans la loi de programmation de la recherche. Quant aux investissements planifiés à l'horizon 2030, ils sont beaucoup trop tardifs pour répondre aux différentes crises climatiques et sanitaires, qui appellent une réaction immédiate.

Depuis 2013, année de création de cette prison, nous en sommes déjà à la sixième prise d'otage selon le même protocole. En 2019, à la suite d'un attentat terroriste islamiste et d'une prise d'otage, j'alertais votre prédécesseur, qui me promettait des moyens supplémentaires pour les gardiens et m'assurait de sa détermination à renforcer la sécurité dans les prisons. Qu'en est-il ? En réalité, deux ans après, rien n'a changé. Les violences et le mépris constituent le quotidien de nos gardiens. toujours autant d'armes artisanales et de téléphones qui circulent sans que les agents puissent fouiller systématiquement les détenus et les visiteurs. Hier, vous vous êtes déplacé pour rencontrer les surveillants. Voici ce que vous avez déclaré à la presse : « J'ai pu rencontrer la jeune surveillante. Elle est profondément choquée d'avoir vu son collègue avec un poinçon sous la gorge. Avec les psychologues, nous allons tout faire pour l'aider à passer cette épreuve difficile. » J'en conclus que, pour vous, la solution, c'est le psychologue en disant : « J'ai tenu à rencontrer le personnel pénitentiaire. Le personnel a présenté des difficultés et des revendications. Nous allons travailler à toutes ces questions. » Bilan : nos interventions ne servent à rien,

» Voilà la vérité ! Vous avez sans cesse de la compassion pour les détenus, en tout cas plus que pour les gardiens et les victimes ! Je réitère donc ma question de 2019 : quand allez-vous permettre aux gardiens d'effectuer des fouilles systématiques et les équiper de pistolets à impulsion électrique comme ils vous le demandent ?

parfaitement autorisées dans certaines conditions. Pour le reste, je tiens à vous dire qu'un travail est actuellement mené, en lien avec les représentants des personnels, pour renforcer la formation

monsieur le sénateur, vous vous mobilisez, comme d'ailleurs Mme la sénatrice Nathalie Goulet, qui suit ces questions depuis fort longtemps. Je vous annonce également que le budget 2022, si vous le votez, permettra de créer 600 emplois supplémentaires dans l'administration pénitentiaire.

Comme votre prédécesseur, vous vous réfugiez derrière les droits de l'homme et dites que vous ne pouvez rien changer. J'imagine que vous allez oublier ce dossier et le redécouvrir à la prochaine tragédie

Les 24, 25 et 26 septembre 2021, les sages-femmes ont déclenché un mouvement de grève dans plus de 150 maternités et dans plus de 60 % des cabinets libéraux. Une nouvelle mobilisation aura lieu demain, jeudi 7 octobre, pour la sixième fois cette année.

Ces conditions de travail, qui se détériorent sans cesse, mettent à mal la permanence et la qualité des soins. Rappelons que, cet été, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes tirait la sonnette d'alarme le manque d'effectifs dans les maternités ne permettait plus de garantir la sécurité des patientes, et que de nombreuses maternités avaient dû fermer leurs portes. Le 16 septembre, monsieur le ministre, vous avez annoncé une revalorisation financière de 100 euros brut par mois,

Comment améliorer, sans moyens réels, la prise en charge des femmes ? Comment rendre la profession attractive ? Ce déficit d'attractivité sans précédent des maternités est dès lors un enjeu de santé publique majeur. Monsieur le ministre, il est urgent d'entendre l'inquiétude et la colère des sages-femmes. Leurs revendications dépassent la seule défense de leur profession : c'est avant tout les femmes, leur santé physique et mentale et celle des nouveau-nés que les sages-femmes défendent.

La décision de la Commission européenne de mettre en oeuvre ce pacte est une bonne nouvelle, alors que la pression migratoire ne fait que s'accentuer. Je souhaiterais vous interroger sur une proposition importante, bien qu'absente du projet présenté le 23 septembre 2020. Le pacte prévoit aujourd'hui un filtrage à l'entrée incluant l'identification de toutes les personnes franchissant sans autorisation les frontières de l'Union européenne ou ayant été débarquées après une opération de sauvetage. Cependant, cette approche axée uniquement sur nos frontières risque de rendre inefficace notre volonté de traiter et d'anticiper l'immigration. Le Conseil européen du 29 juin 2018 était parvenu à s'entendre sur un point intéressant la création de plateformes de débarquement en dehors des frontières de l'Union européenne. Il s'agit d'examiner les demandes d'asile dans des centres gérés et financés par les pays européens.

Bien sûr, il faut convaincre les pays de départ de l'intérêt d'une telle coopération, ainsi que ceux où se situent les principaux points de passage, mais une action coordonnée des instances européennes et des États membres nous permettrait d'obtenir la force d'entraînement nécessaire. Madame la ministre, la France va-t-elle enfin agir pour traduire la proposition du Conseil européen de juin 2018 en actes ? Va-t-elle se mobiliser pour rendre effectif un traitement de l'immigration qui nous permettra de ne plus subir ces flux et empêchera les drames humains ?

depuis janvier, ces professionnels sont déjà descendus plusieurs fois dans la rue pour réclamer davantage de reconnaissance, que ce soit par le biais d'une revalorisation salariale- on vient d'en parler -ou par une augmentation des effectifs dans les maternités. À la suite des premières mobilisations, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles et vous-même avez confié une mission à l'IGAS sur l'évolution de la profession de sage-femme. En effet, malgré toutes les compétences requises et les tâches assumées, les sages-femmes ont aujourd'hui le sentiment de ne pas être reconnues à la juste valeur du travail effectué. Pis encore, elles ont parfois l'impression d'être « maltraitantes » faute de pouvoir accorder le temps nécessaire à chaque patiente. Cette situation s'explique aussi par une pénurie criante de gynécologues dans les hôpitaux. Elles le disent toutes, monsieur le ministre : les sages-femmes ont à coeur de s'occuper au mieux des patientes. Vous avez déjà formulé plusieurs propositions pour la profession.

Des dirigeants d'établissement privé m'ont interpellé à ce sujet, et j'imagine aisément qu'ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la situation. Monsieur le ministre, quelles autres réponses allez-vous apporter pour traiter ces iniquités et répondre aux demandes légitimes de cette belle profession ?

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui vient de publier une circulaire censée répondre à la situation des élèves transgenres dans le milieu scolaire. Il s'agit là d'un sujet grave, que je regrette de voir traiter ainsi avec tant de légèreté. S'il est un fait que la société doit prendre en compte des situations d'élèves ou de jeunes confrontés à ce que l'on appelle désormais une dysphorie de genre, cette circulaire place désormais les directeurs d'établissement et les personnels enseignants en charge d'instituer une nouvelle identité de genre choisi par l'élève à partir de son seul ressenti intime, ce qui se traduit, entre autres, par un changement de prénom. Est-ce bien de la responsabilité des équipes enseignantes d'être, à la fois, officiers de l'état civil, de fait, pour officialiser une identité d'usage, et gendarmes en charge de faire respecter cette nouvelle identité au sein de leur établissement ? Oui ! Sous peine de quelle sanction, d'ailleurs ? La responsabilité de l'équipe éducative consiste à écouter, orienter et protéger les élèves. Mais est-ce bien le rôle des enseignants de les accompagner dans une transition identitaire individuelle et de l'opérer en première ligne, comme préconisé par M. le ministre, avec une médiation avec les familles pour favoriser cette transition ?

S'il est légitime de prendre en considération ces situations quand elles existent, et de leur apporter une réponse adaptée et individualisée, l'approche de ce texte est tout autre. M. le ministre demande, par exemple, le changement des règlements intérieurs sur les tenues vestimentaires pour faire des exceptions la règle.

monsieur le ministre, l'école est-elle encore ce sanctuaire au sein duquel on protège les élèves des excès et des violences de la société, comme des discours militants ?

et de tous est évidemment indispensable pour créer des environnements scolaires propices, favorables et garantissant le droit des élèves à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité. Avec Jean-Michel Blanquer,

et accompagner les situations individuelles, comme vous l'avez dit, et des éléments pour bâtir une politique de prévention de la transphobie à l'échelle de l'établissement scolaire.

ces territoires opaques du monde financier. Alors que d'aucuns dissertent doctement sur l'idée de travailler jusqu'à 67 ans- pourquoi pas 80, tant qu'on y est

Nous devons sortir du mythe selon lequel le système offshore est un outil neutre, simplement mal utilisé par certains. En lui-même, ce système est porteur d'inégalités, car il permet de rompre le contrat social et pousse les plus riches à faire sécession. Certains sur ces travées étaient bien plus prolixes quand il s'est agi d'aborder le séparatisme religieux ; leurs voix se font moins sonores lorsque ce séparatisme se fait financier. Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous sortirez prochainement de ce silence assourdissant. Pas d'« argent magique », donc, pour les services publics, mais beaucoup d'argent caché au service des plus riches. Les écrans plats ! Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner clairement les mesures que vous comptez mettre en place afin d'arrêter cette hémorragie que constitue la fuite des capitaux français dans des paradis fiscaux ?

Au niveau européen, les échanges de données, portant sur 84 millions de comptes et concernant plusieurs milliers de milliards d'euros d'actifs, ont permis à l'Europe de détecter des fraudes et d'encaisser plus de 100 milliards d'euros de revenus complémentaires. Nous avons mis en place des systèmes nouveaux, y compris d'information. Nous avons par exemple pérennisé le système de la rémunération des aviseurs, système proposé par votre collègue de l'Assemblée nationale, Christine Pires Beaune.

en première année de médecine à Paris ont eu une vingtaine de minutes pour préparer un oral sur des thèmes aussi variés que le racisme ou les barrières de corail. L'idée était de diversifier les profils des futurs soignants, en leur posant des questions de société ... Admettons ! Mais le résultat est qu'une quarantaine d'étudiants, en tête des classements à l'écrit, n'ont pas dû avoir des avis suffisamment éclairés sur la vie sous-marine. Cet oral, qui comptait pour 70 % de leur note finale, les a déclassés, barrant ainsi leur passage en seconde année, sans possibilité de redoubler.

au profit des révisions. Je partage totalement le sentiment de ces étudiants d'avoir été volés. Madame la ministre, que comptez-vous faire aujourd'hui pour ces étudiants sacrifiés ?

entament ou poursuivent leurs études de santé. Je veux leur dire à quel point leur présence a été importante durant la pandémie que nous venons de vivre.

que l'année dernière. Pour répondre précisément à votre question, monsieur le sénateur Houpert, personne ici ne souhaiterait que les jurys de concours soient menés par les politiques. Les épreuves que vous évoquez ont été pensées

Lors de son déplacement en Polynésie française, à la fin du mois de juillet, le Président de la République a déclaré à propos du développement des parcs éoliens : « Là où ils créent trop de tensions, dénaturent et défigurent le paysage, il faut savoir ou les adapter ou y renoncer. » Je saisis l'occasion de cette déclaration pour attirer l'attention sur le parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc. Ce parc est d'abord un projet mal né. Sans prise en compte des particularités des fonds marins, sans étude d'impact sérieuse et sans véritable concertation avec les principaux utilisateurs- les pêcheurs -de l'espace maritime concerné, il est effectivement en passe de faire l'unanimité contre lui. Il apparaît clairement que les travaux nécessaires à son implantation provoquent la destruction des fonds marins. Ces désordres, préjudiciables à la biodiversité, vont impacter directement les activités de la pêche côtière et, par conséquent, le gisement de coquilles Saint-Jacques de la baie. Par ailleurs, défigurer le paysage du cap Fréhel, classé au titre des grands sites de France, en implantant 62 éoliennes de 207 mètres de haut à 15 kilomètres des côtes, serait un non-sens. Pour mémoire, la tour Montparnasse mesure 210 mètres. Que les choses soient claires, mesdames, messieurs les ministres : les énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore, doivent être développées en complément de notre production nucléaire, mais pas n'importe où, pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix quel prix ! Compte tenu des propos du Président de la République, le Gouvernement serait-il prêt à renoncer à ce projet et à réfléchir à une ambition alternative plus réaliste et plus adaptée aux caractéristiques de nos côtes ? qui a la particularité d'être implanté plus loin des côtes et ne nécessite pas de forages profonds. Cerise sur le gâteau, le Conseil d'État ayant relevé des irrégularités, le parquet national financier vient de se saisir du dossier d'attribution de ce marché à Iberdrola. Sans commentaire

et, dans ce contexte, pour garantir l'approvisionnement électrique des Français, nous devons développer massivement les énergies renouvelables, dont l'éolien terrestre et maritime. Notre pays dispose du deuxième gisement potentiel d'Europe pour l'éolien en mer. Cette source d'énergie, durable, sûre, compétitive

et dans son exploitation. Comme vous, monsieur le sénateur Cadec, nous avons été très sensibles à l'incident qui s'est produit cet été. Il s'avère que, quand nous avons caractérisé ces huiles, elles se sont révélées biodégradables, selon les normes classiques. Il n'est pourtant pas question, évidemment, de voir de tels incidents se reproduire

La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jacques Bellanger, qui fut sénateur des Yvelines de 1986 à 1995 et de 1997 à 2004. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à permettre l'examen par le Parlement de la ratification de l'ordonnance n° 2021-702 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, présentée par MM. Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, Guillaume Gontard, Jean-Pierre Sueur et François Noël Buffet Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente,

Il va plus loin en explicitant : la démocratie, c'est rendre la parole au peuple. Son propos est sans ambiguïté. Refonder la République, c'est remettre sur pied l'administration autour du Gouvernement, à Paris, mais aussi localement.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons cette après-midi la proposition de loi tendant à permettre l'examen par le Parlement de la ratification de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État. Cette ordonnance remanie en profondeur la conception française de la haute fonction publique de l'État, héritée de l'ordonnance du 9 octobre 1945, prise par le général de Gaulle. Si elle a connu depuis lors des aménagements dans son fonctionnement, la haute fonction publique française, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'en demeure pas moins structurée par un certain nombre de principes fondamentaux, parmi lesquels figurent l'affirmation du primat d'une fonction publique de carrière, la logique de corps, ou encore l'indépendance des fonctions juridictionnelles et des inspections générales. En remettant en cause lesdits principes, cette ordonnance procède à un changement de paradigme majeur ; au travers de ses dispositions, c'est bien le fonctionnement de l'État lui-même qui est en jeu. C'est dire combien le débat que nous nous apprêtons à consacrer à cette réforme est essentiel. Pourtant, il aurait bien pu ne jamais avoir lieu. En effet, non seulement le Gouvernement a choisi de mener cette réforme par voie d'ordonnance, mais il n'a pas montré d'empressement particulier à inscrire son projet de loi de ratification à l'ordre du jour du Parlement.

! Aussi, il faut savoir gré aux présidents Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille et Guillaume Gontard, au président de la commission des lois, François-Noël Buffet, et à notre collègue Jean-Pierre Sueur d'avoir déposé cette proposition de loi. Le présent texte nous permet aujourd'hui d'ouvrir le débat parlementaire sur le bien-fondé des mesures prises dans ce cadre. Comme vous le Comme vous le savez, cette ordonnance traduit l'engagement de l'exécutif à réformer la haute fonction publique de l'État. Elle vient avant tout concrétiser l'annonce phare du Président de la République : la suppression de l'École nationale d'administration et du système dit « des grands corps ». Elle s'inspire en partie du rapport de la mission Thiriez, remis en février 2020.

Il a préféré proposer une nouvelle rédaction, plus encadrée. Si l'article 59 a ouvert un large champ d'habilitation, les garde-fous qu'il comporte- la garantie du principe d'égal accès aux emplois publics, fondé « sur les capacités et le mérite », ainsi que la prise en compte « des spécificités des fonctions juridictionnelles » -sont largement issus de la rédaction adoptée par le Sénat. Comprenant seize articles, l'ordonnance a trois objectifs principaux dynamiser les parcours de carrière de l'encadrement supérieur ; ensuite, rénover la formation initiale et continue ; enfin, décloisonner la haute fonction publique de l'État. Je n'évoquerai qu'une partie de ces dispositions. d'administration (ENA), l'article 5 crée l'Institut national du service public (INSP), qui formera les administrateurs de l'État. Ce nouveau corps constituera le corps unique de sortie de l'INSP, là où les élèves de l'ENA sont actuellement affectés dans dix corps distincts. la répartition des élèves à la sortie de l'ENA est bien moins éclatée qu'il n'y paraît : les administrateurs civils, corps interministériel par excellence, constituent en effet le premier corps de sortie, avec plus de la moitié des affectations. En parallèle, les corps du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des trois inspections générales réunis regroupent moins d'un quart des postes de sortie- je ferme ici cette parenthèse. Que deviendront les actuels corps de hauts fonctionnaires dans la réforme voulue par le Gouvernement ? le Gouvernement ? Si les statuts des corps de fonctionnaires autres que juridictionnels relèvent de la seule compétence du pouvoir réglementaire, certaines dispositions législatives de l'ordonnance ouvrent la voie à la fonctionnalisation d'une grande partie des emplois de la haute fonction publique de l'État. Il en va ainsi des inspections générales : en vertu de l'article 6 de l'ordonnance, les emplois au sein des services d'inspection générale seront désormais occupés par des agents recrutés, nommés et affectés pour une durée renouvelable. L'article 10 permet quant à lui une généralisation des statuts d'emplois, qui pourront déroger à certaines dispositions du statut général de la fonction publique. Bon nombre de postes pourraient être concernés, des fonctions diplomatiques aux fonctions préfectorales. Les juridictions administratives et financières se voient quant à elles réserver un traitement distinct, imposé par des exigences constitutionnelles et conventionnelles. L'ordonnance n'en prévoit pas moins de nouvelles modalités d'accès et de déroulement de carrière pour leurs membres. Le Conseil d'État et la Cour des comptes conserveront leurs corps respectifs. En revanche, ces derniers ne seront plus accessibles directement à l'issue de la scolarité, mais uniquement après une première expérience comme administrateur de l'État. Le grade d'auditeur dans ces juridictions sera remplacé par un statut d'emploi d'une durée maximale de trois ans. Un comité consultatif sélectionnera les candidats, tandis que l'entrée dans le corps sera soumise à l'avis d'une commission d'intégration.

l'ordonnance ouvre aux agents contractuels les fonctions juridictionnelles de maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État et de conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes, ainsi que les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes.

seul le décret fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'État et à la Cour des comptes a été publié à ce jour. Madame la ministre, d'après le calendrier indiqué par votre cabinet, ce chantier réglementaire devrait aboutir au cours du premier trimestre de 2022. Dans ces conditions, la commission a jugé difficile de se prononcer sur des dispositions d'une portée incertaine. Certains contours de la réforme se précisent d'ailleurs au gré des annonces gouvernementales : ainsi, nous avons appris la semaine dernière que les principes de la réforme seraient appliqués à l'ensemble des inspections générales générales actuellement constituées en corps, et non pas seulement aux inspections générales accessibles à la sortie de l'ENA. Au-delà de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales,

l'iceberg. Pouvons-nous nous contenter, en la ratifiant, de donner maintenant un blanc-seing au Gouvernement pour attendre patiemment qu'il précise la portée de la réforme envisagée ? Je ne le pense pas. pas. À cette incertitude réglementaire s'ajoute une incertitude d'ordre jurisprudentiel. Madame la ministre, vous n'êtes pas sans savoir que cette ordonnance n'a pas laissé indifférents un certain nombre de syndicats et d'associations représentant plusieurs corps de la haute fonction publique d'État. l'été, elle a fait l'objet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité auprès du Conseil d'État. Lors de l'audience du 20 septembre dernier, le rapporteur public a recommandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une partie de ces questions ; mais, pour l'heure, le Conseil d'État n'a pas encore statué sur ce renvoi.

En revanche, nous souhaitons que son examen cette après-midi soit l'occasion d'un vrai débat : il n'est pas tolérable que le Parlement soit mis à l'écart, face à des enjeux si importants pour la haute fonction publique de l'État, pour le fonctionnement de l'État lui-même et pour le lien de confiance qui doit unir l'État aux Français.

pris : « Le statut des fonctionnaires ne sera pas remis en cause, mais il sera modernisé et décloisonné, par un assouplissement du système rigide des corps. Nous mettrons en particulier fin au système des grands corps ». Ne vous déplaise, cette réforme était donc une promesse faite aux Français. Depuis 2017, le Gouvernement, avec le soutien de la majorité, a conduit avec détermination cette réforme ambitieuse de notre fonction publique.

En 1945, notre pays sortait exsangue d'une guerre qui commandait de tout reconstruire. Le général de Gaulle engageait alors une refonte sans précédent de nos institutions et de notre administration. La refondation de la haute fonction publique était au coeur de ce projet de restauration de l'État. Ainsi furent créés par ordonnance, non sans résistance à l'époque, l'École nationale d'administration et le corps des administrateurs civils.

Aujourd'hui, notre pays fait face à des besoins nouveaux, ... Bien sûr ! ... radicalement différents de ceux de 1945 : bouleversements technologiques, choc climatique, crises sanitaires, besoin réaffirmé de proximité, etc. La France du XXI siècle, n'est plus celle de 1945, et l'État doit donc de nouveau s'adapter. En dépit de cet impératif, l'État s'est rigidifié, et sa haute fonction publique avec lui : les corporatismes se sont renforcés.

Combien de gouvernements avant nous ont promis de s'atteler à cette réforme de la haute fonction publique ? Ils ont tous échoué. Aucun ne l'a conduite jusqu'à son terme. Je vous rappelle que la suppression de l'ENA figurait déjà dans le programme commun de 1972. En 1995, le Président Chirac promettait, en parlant du classement de sortie de l'ENA, de mettre fin à « une caste qui se coopte ». son Premier ministre, Alain Juppé, annonçait à son tour qu'il allait supprimer l'ENA. Eh oui ! En 2008, une commission mandatée par le Président Sarkozy promettait d'aboutir à un nouveau mode de recrutement « moderne et transparent » pour nos hauts fonctionnaires. Après les juges, c'est le Sénat qui a fait obstacle

Cette réforme exige de la détermination et de la conviction, tout d'abord pour parler aux Français de ce que nous faisons pour eux, ensuite pour parler aux hauts fonctionnaires de ce que nous faisons pour eux ; pour parler de la transformation profonde de l'État que nous menons.

l'efficacité et l'égalité sont les trois conditions absolues de la restauration de l'autorité de l'État. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons décidé de nous attaquer à la racine du problème. Le premier sujet, c'est la formation. Nous devons changer la formation initiale et continue, pour que nos hauts fonctionnaires comprennent la France dans son intimité et dans sa complexité et pour que nous puissions adapter nos politiques publiques, de les différencier selon les territoires. Nous devons faire en sorte que tous nos hauts fonctionnaires acquièrent une culture commune, pour que les décisions ne soient plus prises en silos- les élus locaux sont les premiers à s'en plaindre et ils ont raison.

après la crise sanitaire, et alors que nous devons relever le défi de la relance, c'est bien dans ces ministères et dans leurs services déconcentrés que nous avons besoin de nos nouveaux hauts fonctionnaires. Vous parliez de confiance, monsieur Retailleau. Pour que les Français fassent confiance à l'État, ils doivent voir que l'État s'organise, s'adapte et se soucie des enjeux prioritaires de son époque.

Permettez-moi de vous dire que je considère pour le moins étonnant d'inscrire à l'ordre du jour votre propre texte, afin de le rejeter purement et simplement. du jour la ratification d'une ordonnance pour ne pas la ratifier, je dois dire que c'est assez inédit dans les annales parlementaires ! C'est votre

Que devons-nous déduire de ce jeu politique ? Que M. Retailleau et M. Sueur ne se sont peut-être pas entendus pour déposer des amendements communs ? Que vous ne partagez pas la même vision de l'État ?

Je reconnais bien là les conservatismes de tous bords dont je ne partage évidemment pas la vision. Je reconnais bien là une alliance contre-nature sur plusieurs travées, sans cohérence, sans vision, qui n'a pour objet qu'une opposition stérile et complète au Gouvernement. Les Républicains, les socialistes, les écologistes et les centristes semblent s'accorder, au fond, sur une seule chose : il ne faudrait rien changer.

Il m'avait pourtant semblé avoir lu et entendu des propositions relatives à la fonction publique, formulées notamment à la droite de cet hémicycle. Dans le programme du parti Les Républicains, rendu public ces derniers jours, il est écrit en toutes lettres, monsieur Retailleau, que vous comptez supprimer le statut de la fonction publique et conserver les grands corps-

à laquelle plus de 7 300 d'entre eux ont répondu- exercice absolument sans précédent, que j'ai tenu à mener, visant à nous assurer de la cohérence des décisions que nous prenions avec leurs attentes.

Je regrette le choix qui a été le vôtre de consacrer ce temps parlementaire précieux à un débat par définition stérile, qui se résume à une opposition de principe. C'est sûr ! Soyez assurés de la détermination qui est la mienne, sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre,

contre les corporatismes, contre les immobilismes, pour les agents publics, pour l'État, pour la France et pour les Français. C'est la raison pour laquelle je donnerai bien sûr un avis favorable à cette proposition de loi, qui propose la ratification d'une ordonnance posant les jalons de la réforme de notre haute fonction publique la plus ambitieuse depuis 1945. Je suis saisie,

par sa famille, par des relations ou par tel ou tel réseau. C'est extrêmement grave ! Vous faites le contraire de ce que vous dites. Vous faites quelque chose d'antidémocratique et vous mettez à bas en définitive toute la réforme de la fonction publique de 1945. Jusqu'à présent, le personnel de la fonction publique a toujours été géré en fonction du mérite et des capacités de chacun, appréciés sur la base d'éléments objectifs. Ainsi, les nominations et les promotions dépendent de la valeur personnelle et de la réussite aux concours et examens- y compris pendant toute la carrière, car il existe des concours internes -et non d'appréciations subjectives. Le système, à défaut d'être parfait, est au moins juste. Or, sous couvert d'une fausse égalité des chances, le Gouvernement veut remplacer ce système par une logique de nominations au jour le jour, en fonction d'appréciations totalement subjectives et arbitraires. Cela permettra de généraliser un favoritisme systématique et profondément injuste. C'est déjà le cas actuellement pour la nomination de certains préfets à des fonctions n'ayant rien à voir avec l'administration préfectorale, ou pour certains ambassadeurs. Citons

La carrière d'un fonctionnaire doit dépendre de sa valeur. Hélas, avec le système qui sera mis en place, ceux qui réussiront sont ceux qui ont des relations familiales, ceux qui font partie de réseaux occultes- par exemple, la franc-maçonnerie

Madame la ministre, lors des questions au Gouvernement du 9 septembre 2021, je vous ai posé la question suivante, que je reprends mot pour mot. La carrière des fonctionnaires était jusqu'à présent organisée sur des bases claires, tenant compte de leur réussite aux concours et aux examens. Elle dépendait donc de critères objectifs. À défaut d'être parfait, ce système était au moins juste. d'une fausse égalité des chances, le Gouvernement veut le remplacer par des nominations et des promotions au jour le jour, fondées sur des appréciations qui seront inévitablement arbitraires. Cela conduira inéluctablement à des passe-droits.

C'est ce que je vous ai dit. Vous avez très bien compris, lorsque j'ai posé cette question, que je défendais les hauts fonctionnaires et la fonction publique en général, dans sa configuration issue de la loi de 1945.

Pis, vous avez tenu à mon égard des propos désobligeants et d'une totale mauvaise foi, comme vous l'avez fait à l'encontre de M. Retailleau tout à l'heure ! Pauvre victime ... Vous avez prétendu que je critiquais la compétence et le travail des fonctionnaires, alors que j'avais dit exactement le contraire. Je cite vos propos, madame la ministre : « Ministre de la fonction publique, je ne saurais laisser passer qu'à coups de complotisme ou de vous remettiez en cause la compétence et l'engagement de ses hauts fonctionnaires.

singulier. Comme l'a souligné Mme la rapporteure, dont je salue le travail, nous ouvrons la première discussion parlementaire d'une proposition de loi de ratification d'une ordonnance. C'est la première fois fois que cela se produit. Néanmoins, ce qui est singulier, c'est surtout que les auteurs de cette proposition de loi voteront tout à l'heure, comme ils l'ont fait en commission, contre le texte qu'ils ont eux-mêmes écrit et dont ils ont souhaité l'inscription à l'ordre du jour de notre assemblée. Avouez que c'est assez surprenant et paradoxal processus est inédit, bien qu'il soit attendu dans son aboutissement. En fait, ce rejet vous permet, mes chers collègues, d'afficher une opposition ferme et entière à la réforme de l'encadrement supérieur de l'État conduite par le Gouvernement. Cela, nous l'avons bien compris. là encore, admettez que l'on peut s'étonner d'un rejet délibéré et en bloc d'une proposition de loi dont la force était justement d'ouvrir à toutes sortes de modifications l'ensemble des dispositions de l'ordonnance contestée sur ces travées, le véhicule de nos collègues se trouvant finalement limité par ses propres auteurs à un moyen de débat, à rebours du vecteur de propositions et de solutions de rechange de fond qu'il aurait pu être. Dont Au-delà de ce choix innovant, et même disruptif, si j'ose dire, de la majorité vastement élargie de notre assemblée, plusieurs points pouvaient nous rapprocher. Déjà, nous ne contestons pas le principe ni l'initiative d'inscription d'une proposition de loi de ratification à l'ordre du jour de notre Haute Assemblée. Je vous l'ai dit. Il est tout à fait loisible au législateur d'y procéder, dès lors que, passé le délai d'habilitation, seule la loi peut modifier l'ordonnance, et dès lors, aussi, qu'une telle inscription garantit la tenue au Parlement d'un débat sur la réforme de la haute fonction publique de l'État. permet au Gouvernement de répondre à des craintes qui doivent être entendues et de faire un état des lieux du vaste chantier réglementaire en cours, qui sera déterminant pour les contours concrets de la réforme. Je pense notamment à la création des statuts d'emplois et aux garanties qui y seront attachées en matière d'indépendance, mais également de compétences impliquées par la spécificité de certaines fonctions. Pourtant, le rejet en bloc décidé par nos collègues de la majorité traduit mal la réalité du débat et de ses termes. L'opposition au texte de ratification viserait, pour certains, à fustiger le contenu de la réforme, voire l'idée même d'une réforme de la haute fonction publique, et, pour d'autres, à prendre acte d'une difficulté d'appréciation de l'ordonnance, liée à des procédures pendantes et à un vaste chantier réglementaire en cours. S'agissant de ce dernier argument de l'impossibilité matérielle, permettez-moi de souligner que le calendrier d'examen de la proposition relève d'un choix de la majorité sénatoriale et qu'il peut donc difficilement être imputé à des tiers. Pour ce qui est du rejet en bloc de la réforme, celui-ci ne traduit pas les points de convergence qui auraient pu se dessiner au moins sur les objectifs. Nous aurions pu trouver des objectifs communs. L'idée de réformer la haute fonction publique n'est pas réductible à une lubie d'un président de la République et de son gouvernement, qui se rendraient au chevet des passions tristes d'une partie de la société en s'attaquant à l'élitisme et au modèle français

En effet, plusieurs objectifs de la réforme pourraient autoriser une certaine convergence de vue de plusieurs groupes. Je pense, bien sûr, au renforcement de l'interministérialité, dans la continuité de l'ordonnance de 1945 de ses motifs d'une « spécialisation et [d']un cloisonnement excessifs » des administrations. Pour affermir cette interministérialité, l'ordonnance du 2 juin 2021 décloisonne la haute fonction publique en renforçant les mobilités et en mettant fin au déterminisme du classement de sortie. Elle dynamise les parcours de carrière de l'encadrement supérieur, en mettant en place une gestion des ressources humaines plus stratégique, interministérielle et, surtout, davantage individualisée. Au coeur de cette réforme se loge un autre point sur lequel nous pouvions nous entendre : la meilleure valorisation des fonctions opérationnelles, par les exigences de mobilité, et les conditions d'accès posées pour certains corps et certains grades- en cohérence avec l'idée, que je partage bien volontiers, du terrain comme première compétence, comme niveau où les décisions concrètes doivent être prises. Je soulignerai pour terminer la dissonance entre le rejet en bloc qui nous est proposé cette après-midi et le rapport du Sénat sur la loi de 2019 de transformation de la fonction publique, dans lequel étaient défendus les objectifs suivants, qu'il me semble retrouver dans la présente réforme : la création d'un tronc commun d'enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines la prise en compte des expériences professionnelles et de la connaissance des territoires ; enfin, le développement de la formation continue des agents et la meilleure gestion de leurs parcours de carrière. Voilà des thèmes qui nous étaient communs, que nous pouvions défendre, mais qu'aucun d'entre vous n'a repris.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aborde deux sujets importants. Malheureusement, elle apporte une réponse incompréhensible. Le premier sujet concerne les ordonnances. Depuis des décennies, sous ce gouvernement comme sous les précédents, nombre d'entre elles ne sont pas ratifiées, et elles le sont de moins en moins. Une fois l'habilitation votée, le Parlement perd la maîtrise des dispositions qui sont décidées par l'exécutif. Le défaut de ratification n'entraîne pas, en l'état de la jurisprudence constitutionnelle, la caducité de l'ordonnance. Le seul dépôt du projet de loi de ratification suffit à sa validité. Cet état de fait incite évidemment le Gouvernement à se passer de l'avis du Parlement sur un certain nombre de textes. Cette méthode est condamnable, parce qu'elle constitue un contournement de l'esprit de la procédure d'habilitation à légiférer par ordonnances. Alors que l'article 38 de la Constitution dispose qu'une ordonnance ne peut être ratifiée que de manière expresse, la pratique se dispense d'une telle ratification. Cet entre-deux n'est pas satisfaisant, et cette PPL a le mérite de poser le problème. second sujet abordé par ce texte est celui du fond de cette réforme. Il y a longtemps qu'elle était souhaitée et envisagée par la droite et le centre. Les nécessités d'ouvrir la haute fonction publique, d'ancrer les carrières dans les territoires, de réformer l'ENA, de lutter contre le déterminisme ne datent en effet pas d'hier. En 2008, le président Sarkozy jugeait déjà « choquant » que « le résultat d'un concours passé à 25 ans oriente toute une vie professionnelle ». Il a tenté à plusieurs reprises de supprimer le classement de sortie de l'ENA, sans y parvenir. Aujourd'hui, le Gouvernement réalise la réforme que la droite et le centre appelaient de leurs voeux. Les fonctionnaires issus du futur Institut national du service public devront tous se confronter à la réalité du terrain, en occupant des fonctions opérationnelles. Cette expérience est indispensable pour pouvoir conseiller ou juger les politiques menées par l'État. La mobilité est également incontournable pour connaître les postes de celles et ceux que l'on sera amené à encadrer. Enfin, il est sain que les carrières de nos hauts fonctionnaires évoluent en fonction des résultats de l'évaluation de leur action. Cette réforme n'est peut-être pas parfaite, elle ne va peut-être pas assez loin, mais elle va déjà bien plus loin que quiconque ne l'a fait depuis 1945. Dans leur démarche contre la réforme proposée et pour la procédure de ratification, les auteurs de cette PPL se sont tiré une balle dans chaque pied, et une troisième on ne sait où, puisqu'il n'y a que deux pieds Première balle dans le pied : le Parlement peut toujours modifier les dispositions d'une ordonnance à l'expiration du délai d'habilitation. Pourquoi ne pas avoir amendé le texte de l'ordonnance et voté sur un texte amélioré par le Sénat, plutôt que de voter contre le propre texte que l'on dépose ? Évidemment, il aurait fallu que les quatre groupes soient d'accord sur la réforme et les amendements à proposer, ce qui semble bien plus compliqué que de censurer le texte du Gouvernement. Deuxième balle dans le pied : qui, parmi nos concitoyens, comprendra que l'on dépose une proposition de loi de ratification dans le but de rejeter cette même proposition ? Cette démarche est inédite. Elle figurera peut-être un jour dans un recueil des moments savoureux du Sénat ! Troisième balle, qui a certainement rejoint l'une des deux autres le texte de ratification amendant l'ordonnance aurait pu continuer son cheminement parlementaire en portant les modifications du Sénat. Mais, en votant contre son adoption, notre chambre enterre cette possibilité au moment même où elle la rend possible. Pas du tout ! Si ! Comprenne qui pourra. Notre groupe soutient les ambitions de la réforme de la haute fonction publique proposée par cette ordonnance. C'est d'ailleurs aussi le cas des deux groupes de droite qui présentent cette PPL, puisque, en habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance, ils montraient bien qu'ils allaient dans le sens de cette réforme. Parce qu'il s'agit d'une réforme longtemps attendue, nous allons rester logiques avec nous-mêmes. En remerciant les auteurs de ce texte de nous en donner l'occasion, mais contrairement à leurs recommandations, notre groupe votera donc en faveur de cette PPL, en regrettant, hélas, qu'elle soit mort-née.

vous me permettrez tout d'abord de vous dire que nous avons modérément goûté le ton et le contenu des propos que vous avez tenus à l'égard du Sénat dans de ce matin. Je n'ai pas non plus beaucoup apprécié la manière très polémique dont vous avez abordé le débat.

il me semblait que la recherche de terrains d'entente entre la droite et la gauche était au fondement même du macronisme. Par conséquent, je ne vois pas ce qui vous choque dans le fait que plusieurs présidents et membres de groupes différents se soient associés pour obtenir l'inscription de la ratification de votre ordonnance à l'ordre du jour du Sénat.

de la Constitution et constitue une légitimation que vous ne pouvez pas obtenir par une simple signature des membres de l'exécutif.

l'on rejette un texte, parce qu'on le juge non amendable et que l'on refuse de s'inscrire dans les dispositions qu'il prévoit.. Pas quand de votre ordonnance. Je comprends que cela vous contrarie, mais c'est la nature même du débat démocratique que d'échanger des convictions ; les nôtres sont différentes des vôtres, admettez-le, s'il vous plaît.

et de l'esprit de la Constitution. La seconde touche au fonctionnement de l'État, dans le respect de nos traditions républicaines, avec pour seul impératif- je sais que vous le partagez et je n'attaque pas votre bonne foi -, la qualité du service public. Nous empruntons des chemins différents pour atteindre ce second objectif. Ces deux difficultés sont graves et nous conduisent à rejeter votre ordonnance, en formant le voeu que l'Assemblée nationale en débatte à son tour ; cela dépend naturellement de vous, mais aussi des groupes

et vous devez comprendre que nous, représentants de la Nation, en soyons extrêmement irrités. En ce qui concerne

». Vous voyez le niveau auquel se situe le pouvoir d'habilitation du Parlement : il s'agit de choses essentielles. Au fil des années, et pas seulement d'ailleurs sous cette mandature, on a vu se dégrader le niveau d'exigence des lois d'habilitation au regard de la politique générale du Gouvernement, mais je ne conteste pas, après tout, que la réforme de la haute fonction publique de l'État puisse faire l'objet d'ordonnances quand elle est au coeur du programme du Gouvernement. J'observe simplement que

plus on fait de lois, plus on fait aussi d'ordonnances. Nous assistons donc à une saturation de l'action publique par la loi ; tout se passe comme si la fin ultime de toute action du Gouvernement était de légiférer. Notre pays est dans une confusion croissante.

Je ne considère pas que rebaptiser l'ENA « INSP » et y adjoindre les formations pour d'autres catégories de fonctionnaires constitue un réel progrès ; je ne vois pas, au moment où nous parlons de l'amélioration de la prise en compte des métiers, pourquoi il faudrait fondre dans un grand magma toutes les formations des hauts fonctionnaires. Vous avez fragilisé, non pas des corps, mais des institutions constitutionnelles, en modifiant les modalités du recrutement et en les fondant non pas sur le mérite intellectuel, mais sur la pratique administrative. Sachez que, à la Cour des comptes et au Conseil d'État, les qualités opérationnelles ne sont pas les premières qui sont nécessaires pour réussir à maîtriser les outils et les concepts intellectuels mis en oeuvre dans ces institutions constitutionnelles.

durable. Je voudrais vous signaler enfin que votre ordonnance- ce n'est pas son moindre défaut -, dans ses premiers articles, relève purement et simplement de l'instruction du Premier ministre. Voilà une ordonnance qui traite de sujets qui relèvent de circulaires ! Oui, il faut une gestion prévisionnelle des emplois, mais cela n'a pas à figurer dans une ordonnance.

dans des proportions sans commune mesure avec ce que la V République avait connu jusqu'à présent. Votre absence de considération pour le pouvoir législatif ne semble pas connaître de limite. Nous nous retrouvons donc dans une position invraisemblable : nous devons nous autosaisir de la ratification de vos ordonnances pour provoquer le débat parlementaire. S'agissant du sujet qui nous occupe, la réforme de la haute fonction publique, rien, absolument rien ne justifiait le recours à l'ordonnance pour nombre d'articles, ni l'urgence, totalement absente, ni la technicité du sujet. Transformer la haute administration pour l'adapter aux enjeux du XXI siècle, réformer l'ENA et les grands corps, cela nécessitait un débat politique digne de ce nom devant la représentation nationale. Madame la ministre, ne faites donc pas semblant de ne pas comprendre notre démarche commune. Il y aurait Il y aurait beaucoup à dire. Si nous réprouvions la loi de transformation de la fonction publique de juin 2019, qui affaiblissait le statut de fonctionnaire et ouvrait grande la porte des emplois publics à des contractuels recrutés en dehors des concours, souvent dans des conditions précaires, cette ordonnance, qui en émane, n'est pas à rejeter en bloc. La réforme de l'ENA, transformée en Institut national du service public, était nécessaire. L'intégration systématique des grands corps d'État pour les élèves arrivés en tête du classement de sortie était une pratique d'un autre temps un symbole fort de la déconnexion croissante entre les élites politico-administratives et la population, dans notre État jacobin, dans lequel ces administrations sont concentrées dans la capitale., rendre rendre obligatoire pour les futurs diplômés un exercice de cinq années dans les services déconcentrés de l'État est une très bonne mesure. La création d'un corps unique des administrateurs de l'État laisse également espérer plus de mobilité des hauts fonctionnaires au sein de la sphère publique, ainsi que des carrières plus cantonnées à un seul ministère, choisi pour quarante ans dès la sortie de l'ENA. Inclure dans la formation des administrateurs des modules relatifs à la transition écologique, à la transformation numérique de nos économies ou encore aux enjeux de la pauvreté relève du bon sens. « Enfin ! », pourrions-nous dire. Nous n'avons néanmoins pas beaucoup d'illusions sur les évolutions du contenu pédagogique de l'École. Dans une logique néolibérale néolibérale toujours prégnante, on continuera très certainement à y apprendre que la dépense publique est un problème et l'intervention publique dans le secteur économique une hérésie. Nous sommes circonspects sur la suppression du corps des préfets. Nous craignons que cela n'ouvre beaucoup trop les administrations préfectorales à des profils venus du privé. De ce fait, nous nous inquiétons de l'affaiblissement du sens du service public et de l'intérêt général chez les serviteurs de l'État, pour ne pas dire de la multiplication des conflits d'intérêts. C'est bien là que le bât blesse et que nous sommes dans l'incapacité de vous faire confiance. Votre philosophie, exprimée par la loi de 2019, est l'ouverture de la fonction publique et la multiplication des allers-retours entre le public et le privé. Nous nous opposons fermement au pantouflage des grands serviteurs de l'État. Or tout laisse à penser que cette ordonnance, loin de lutter contre ce phénomène délétère, va le favoriser. Ce texte est en effet très général, et l'essentiel de ses dispositions est renvoyé au règlement. L'absence de débat parlementaire est ici préjudiciable, tant il aurait permis d'encadrer le travail réglementaire du Gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre la ratification de cette ordonnance nous espérons que l'exécutif reviendra devant le Parlement pour présenter une ambitieuse réforme de la haute fonction publique. Plus largement, nous demandons l'organisation d'un débat annuel au Parlement sur la gestion des ressources humaines de l'État. Cela doit faire partie de notre mission de contrôle. Pour conclure, il y a quinze jours, le collectif Nos services publics publiait une enquête dans laquelle 80 % des agents interrogés se déclaraient « confrontés à un sentiment d'absurdité dans l'exercice de leur travail

du mandat. Combien de fois avons-nous entendu des ministres, ici même ou plus souvent dans les couloirs ou dans la presse, expliquer que certains hauts fonctionnaires du ministère des finances décidaient

de ce fonctionnaire formé un homme, et non un simple rouage de l'administration. Or ce que vous nous proposez aujourd'hui ne répond en rien

madame la ministre, mes chers collègues, lors de son intervention à l'occasion de la convention managériale de l'État, le 8 avril dernier, le Président de la République a précisé les contours d'une réforme de la haute fonction publique

de l'encadrement supérieur de la fonction publique d'État, que la présente proposition de loi vise à ratifier, concrétise l'engagement présidentiel de réformer la haute fonction publique. Outre l'ENA, l'ENA, elle supprime aussi les grands corps d'État, privilégie les missions opérationnelles pour les premiers emplois, crée des évaluations régulières des pratiques professionnelles et valorise la prise de risques. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 avait habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.

En l'espèce, le Gouvernement a bien déposé un projet de loi de ratification à l'Assemblée nationale le 29 juillet 2021. Toutefois, depuis cette date, rien n'indique qu'il ait l'intention d'inscrire ce texte à l'ordre du jour. l'intention d'inscrire ce texte à l'ordre du jour. Il esquive ainsi le débat parlementaire sur une réforme pourtant substantielle de l'administration. En se saisissant lui-même de la question, le Sénat est à l'origine de la première discussion au Parlement d'une proposition de loi de ratification d'une ordonnance. Une initiative rare, qui

Avant d'évoquer spécifiquement l'ordonnance du 2 juin 2021, le débat de cette après-midi nous offre l'occasion d'évoquer plus généralement l'usage des ordonnances par le Gouvernement depuis plusieurs mois.

Ce recours excessif aux ordonnances vient d'ailleurs d'être dénoncé dans l'étude annuelle du Conseil d'État : « Malgré l'utilité indéniable des ordonnances en période de crise, une utilisation massive accentue fortement le déséquilibre institutionnel au profit du pouvoir exécutif ». Autrement dit, la victime est toujours la même victime : le Parlement ! Pour ne rien arranger, une récente décision du Conseil constitutionnel vient jeter le trouble sur cette question. En effet, dans deux décisions de mai et juillet 2021, le Conseil a reconnu une valeur législative aux ordonnances du Gouvernement non ratifiées par le Parlement, ce qui n'est ce qui n'est pas sans fragiliser le principe constitutionnel selon lequel la loi, expression de la volonté générale, ne peut naître que de la délibération publique. Plus spécifiquement, je rappelle que l'article 38 de la Constitution exige que les ordonnances soient ratifiées de manière expresse. Avec les décisions précitées du Conseil, certains ont évoqué même la création d'une législation par voie gouvernementale. Face à cela, que peut faire le Sénat ? Notre Haute Assemblée est depuis longtemps mobilisée sur ces questions. Nous avons récemment encore été force de proposition, puisque notre règlement vient d'intégrer des outils permettant d'opérer un contrôle plus étroit de la législation déléguée, c'est-à-dire des ordonnances de l'article 38. Nous avons ainsi ajouté le suivi des ordonnances aux missions des différentes commissions permanentes du Sénat et renforcé leur information sur les intentions du Gouvernement quant à leur publication et leur ratification. Voilà pour la forme. Cette proposition de loi ouvre les conditions d'un vrai débat sur l'opportunité et l'intérêt d'une telle réforme. Je rappelle en préambule que, en effet, le Sénat n'a pas émis d'objections à l'habilitation à la mener par voie d'ordonnances en 2019.

Pourquoi supprimer l'ENA pour la remplacer par une autre école, qui ne change ni ses modalités d'accès, ni son classement de sortie, ni même les épreuves du concours externe ? Parler de suppression est d'ailleurs une supercherie : rien n'a été supprimé, On veut faire nous faire croire que l'on a cassé le moule de cette fameuse technocratie qui serait la cause de tous nos maux. Pourquoi supprimer les grands corps de l'État, refuges d'excellence et de méritocratie qui rendaient la haute fonction publique attractive ? Le remplacement des grands corps par un large corps commun interministériel à la gestion centralisée nous garantit-il une meilleure fonction publique ? Certains craignent au contraire une politisation des fonctionnaires, notamment des ambassadeurs et des préfets. Pendant la crise sanitaire, on célébrait tous les matins les vertus du couple maire-préfet, pilier de l'État unitaire décentralisé. Pourquoi aujourd'hui déconstruire un symbole de la République, autour duquel s'est forgée la Nation ? La fonctionnalisation des postes de préfets de département et de région pourrait introduire, demain, le doute sur la qualité de nominations, non plus seulement fondées sur le mérite et l'expérience, mais motivées par la faveur politique.

L'histoire de France est intrinsèquement mêlée à celle des idées politiques, et elle connaît quelques passages incontournables. Parmi ceux-là, je pense aux dernières années de l'Ancien Régime, quand les États généraux venaient d'être convoqués. Il y avait alors une critique presque systématique du mode de prise de décision des gouvernants. Le juriste Guillaume Le Trosne, s'exprimant au sujet de celui qui décidait, qu'il soit Roi, ministre ou administrateur,

ou d'après des rapports infidèles ». Le reproche était assez classique et attendu pour l'époque, la volonté d'un seul homme, même oint du droit divin, ne pouvant plus légitimer une décision. Si je mesure bien la distance historique avec laquelle il faut recevoir cette citation, elle résonne néanmoins par deux fois dans notre discussion d'aujourd'hui. Une première fois au sujet des ordonnances. La tendance à y recourir s'accroît toujours un peu plus et donne le sentiment d'un gouvernement qui entreprendrait « de tout diriger par lui-même », laissant au Parlement le seul soin de l'y habiliter et de n'en contrôler le respect que du bout des lèvres. Sur ce point, les membres du groupe RDSE ont déjà eu l'occasion de le souligner : ils sont réticents par principe au recours aux ordonnances sur des sujets éminemment politiques. Le débat parlementaire doit demeurer l'essence de notre République. Le second point concerne notre haute fonction publique. Les termes du débat qui entouraient la place des intendants, ancêtres des préfets et figures de la monarchie administrative du XVIII siècle, sont finalement assez proches de ceux que nous retrouvons au sujet de nos hauts fonctionnaires, auxquels il est reproché une organisation en corps nettement distincts et trop isolés et dont certaines règles et certains statuts constitueraient des sortes de privilèges perçus comme injustifiables.

qui se substituerait aux représentants de la Nation. L'administration doit demeurer avant tout un outil au service de l'application des décisions des élus, nationaux comme locaux. Je salue donc l'initiative des auteurs de cette proposition de loi. Nous connaissons les problèmes que pose la formation de l'encadrement supérieur. Ils sont identifiés et dénoncés depuis longtemps.

se trouve donc dans les modalités d'organisation de cette formation et dans la concrétisation du nouveau dispositif. En quoi permettra-t-il de former des hauts fonctionnaires qui seront plus en phase avec les territoires plus aptes à comprendre le sens du service public, lorsque celui-ci s'exerce dans sa diversité locale ? En quoi les élèves de ce nouvel institut se démarqueront-ils véritablement des promotions d'énarques ? Les mêmes interrogations planent au-dessus du nouveau corps d'administrateurs de l'État qui aura vocation à accueillir les anciens élèves de l'INSP. L'ordonnance le crée sans le préciser, laissant le soin au seul pouvoir réglementaire d'en décrire les attributions. La logique interministérielle que devra porter ce nouveau métier mérite des éclairages supplémentaires. Au vu de ces différents éléments, nous comprenons très bien les remarques de la commission des lois quant aux incertitudes qui entourent cette ordonnance. Nous comprenons également la demande des auteurs de cette proposition de loi, qui veulent qu'une telle réforme ne se fasse pas sans un vrai débat public. Il reste toutefois assez curieux

l'ordonnance qui nous intéresse transforme en profondeur la conception républicaine que nous avons de la haute fonction publique de l'État, telle qu'elle est issue de l'ordonnance du 9 octobre 1945 et des travaux du Conseil national de la Résistance.

une logique de bouc émissaire, il a tenu sa promesse. Plus encore, l'ordonnance propose de diversifier le mode de recrutement, d'ouvrir la haute fonction publique et de dynamiser la gestion des carrières. Dynamiser », « ouvrir », « diversifier », « flexibiliser », ces mots répétés à l'envi, de manière abusive en ces temps de campagne électorale, perdent de leur force dans l'esprit de nos concitoyens. Les mots lassent. Les actes manquent. Ils manquent pour convaincre que la République mérite encore d'être notre idéal commun, le socle de notre identité. Ces mots sont issus du lexique vaporeux de la « start-up nation » chère au Président de la République. Pour redonner corps à notre République, il faut une action déterminée en faveur de l'égalité.

La méritocratie républicaine rime avec la promesse républicaine. Néanmoins, ne jetons pas un voile pudique sur les concours de la haute fonction publique. Ils se posent comme un modèle suprême d'égalité, mais chacun sait qu'ils ne sont accessibles qu'à un public trié sur le volet,

Réserver quelques places au concours est généreux, mais sans effet structurel. La sélection sociale s'effectue sur le long terme, avec une succession d'entonnoirs. Plutôt que de tenir la promesse d'égalité, le Gouvernement préfère détricoter la haute fonction publique, dans un vase clos.

même de l'indépendance des fonctions juridictionnelles. Le fait du prince, même encadré, deviendra la règle. Madame la ministre, vous n'y pouvez rien, mais votre méconnaissance de l'administration est grande. Vos préjugés culturels sur la nécessité de transposer les méthodes de gestion des cadres dirigeants du secteur privé

Le politique, quand il gouverne, veut paraître moderne. Quoi de plus normal ? Dans votre logique ultralibérale, les fonctionnaires sont des freins et l'administration est inutile. Votre idée est non seulement d'importer les méthodes du privé, mais aussi de réduire les impôts et d'amoindrir l'État, ainsi que ceux qui le servent. fondamentalement, et je le respecte, à la « main invisible » du marché et à son avatar macronien, la théorie du ruissellement. Vous vous trompez de priorité. L'actualité, c'est l'exigence d'un lien entre l'administration et ses administrés et de la connaissance du terrain par les hauts fonctionnaires. Cette préoccupation est unanimement partagée. Comment ne pas voir le fossé qui se creuse entre les citoyens et des hauts fonctionnaires qui se détachent des réalités vécues ? Nous sommes tous d'accord sur ce diagnostic et sur le principe qu'il faut restaurer le lien de confiance qui s'est distendu entre l'État et les Français. Pourtant, la solution n'est ni le délitement de la haute fonction publique ni le remplacement de l'ENA par une ENA . Tout a été dit sur le sujet depuis le début de cette discussion générale. Et en même temps, vous avez pensé que cette remise en cause lourde et structurelle ne méritait pas l'examen de la représentation nationale !

Madame la ministre, vous engagez-vous, au nom du Gouvernement, à ce que l'ordonnance relative à la haute fonction publique adoptée ce matin donne lieu à une ratification explicite, au terme d'un vrai débat parlementaire ? » Vous n'avez pas répondu à la question,

avec nos collègues communistes, lorsque nous nous sommes opposés à cette habilitation, lors de l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique, en 2019. Nous avions proposé, à deux reprises, en commission puis en séance, un amendement de suppression. Cependant, il faut reconnaître

était sous le gouvernement de M. Valls, qui a dû faire face, ne l'oublions pas, aux attaques terroristes. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des ordonnances prises en 2021 pour lutter contre la pandémie.

pour ce gouvernement, tout semble urgent. La procédure accélérée est systématique. Le recours aux ordonnances atteint un niveau record. Les projets de loi déguisés en propositions de loi se multiplient.

La réforme n'aurait-elle pas pu supporter quelques semaines de débat, madame la ministre ? Votre rapport au temps parasite l'activité législative. Vos projets de loi sont de plus en plus réactionnels.

dégrade, je vous le dis très sincèrement, le travail parlementaire, celui de la représentation nationale. Votre rapport au temps se limite à une succession d'instants, sans profondeur historique ni projection dans l'avenir. Vous nous privez de toute négociation sociale et de délibération collective. Vous ne vous projetez pas même à l'horizon d'une génération. Votre nouveau monde est flou, dans un présent perpétuel, indéfini, sans histoire ni utopie, incapable de mettre à distance le contingent. L'utilisation des ordonnances reflète la posture jupitérienne du Président de la République, les dérives d'un pouvoir à bout de souffle, pétri de certitudes, dans un système institutionnel fermé à l'expression citoyenne et à ses représentants. À tenir à distance le Parlement, les corps intermédiaires et le dialogue social, à leur préférer un lien direct avec les Français qui ressemble davantage à une pratique plébiscitaire du pouvoir qu'à un véritable dialogue, vous faites le lit du populisme ; vous comprendrez aisément l'allusion, en cette période d'hypersondages.

Madame la ministre, la France est caractérisée par une administration de grande qualité, loyale et performante. La gestion de la crise sanitaire en a été une nouvelle illustration sur bien des plans. Cette administration est constituée de fonctionnaires qui servent l'État, au sens noble du terme, en exécutant la politique d'un Gouvernement élu démocratiquement et responsable des résultats devant les citoyens. Tel était en tout cas le modèle en vigueur jusqu'à

La réforme de la haute fonction publique, engagée par la mission Thiriez, met l'accent sur quelques travers des corps administratifs : la diversité sociale et académique des recrutements est limitée, la formation continue reste faible, voire inexistante, les carrières sont très dépendantes des résultats au concours de recrutement, le phénomène de « rentes » dans certaines fonctions n'est plus acceptable,

de fonctionnement est souhaitable, à condition de rester une voie complémentaire, il remet en question le modèle d'une fonction publique de carrière, où l'on ne sert pas les intérêts privés, ni avant de prendre son poste, ni en le quittant.

Il s'agit d'un fonctionnaire d'un haut niveau de formation scientifique, pouvant aller jusqu'au doctorat. Il raisonne en projets et non en processus. Il maîtrise un domaine thématique, comme l'armement, la statistique, l'aménagement, l'environnement ou le numérique,

Le modèle promu par l'ordonnance se rapproche du mode de gestion des enseignants. Faudra-t-il bientôt qu'un haut fonctionnaire capitalise un nombre de points pour faire mobilité, comme c'est le cas lorsqu'un enseignant souhaite changer d'académie ? En forçant le trait, voilà ce à quoi pourrait conduire une gestion en masse et non plus individualisée Pour le dire autrement, je ne suis pas convaincue que le modèle d'une fonction publique composée uniquement de fonctionnaires administratifs et d'expertises contractuelles mobilisées à la volée, permette à l'État de mener une politique industrielle, environnementale, d'armement ou d'aménagement qui soit à la hauteur des enjeux auxquels notre pays doit répondre.

Depuis Napoléon, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif. Depuis François I, les ambassadeurs sont nommés par le pouvoir exécutif. La nomination des directeurs d'administration centrale des chefs d'inspection générale - je me tourne vers M. le questeur Bas, qui connaît très bien les procédures de décision et de nomination en conseil des ministres -ne sera pas modifiée : les préfets seront nommés tous les mercredis en conseil des ministres, comme ils l'ont toujours été.

C'est avant tout un engagement à servir un territoire et des projets et à faire travailler ensemble les acteurs publics, les élus territoriaux, les entreprises, bref l'ensemble des acteurs qui font la réussite

Être un patron dans un département ou une région n'oblige pas à être membre d'un corps. Cela oblige, vous l'avez dit, à avoir des compétences, à avoir été formé, à avoir une expérience,

parce que la haute fonction publique et son avenir exigent une loi globale, qui soit l'occasion de clarifier, de débattre et de rendre lisible aux Français ce que l'on fait. En effet, ces derniers n'ont rien compris à votre histoire,

plus votre culture du s'applique pour les hauts fonctionnaires, moins ceux-ci sont en respiration avec la réalité de ce pays, moins ils sont porteurs, dans la durée,

Vous aurez demain des préfets intermittents, intérimaires, fonctionnalisés, contractualisés. Je vois très bien de quoi il s'agit : c'est un système qui met en cause toute une cohérence républicaine,

de vote. Pour ma part, je suis contre l'ordonnance et je n'ai pas voté la loi en question. Indépendamment de cela, rassurez-vous, madame le

monsieur Sueur.

Sénat rejette ce texte, de le soumettre à l'Assemblée nationale. Le Sénat n'avait qu'à assumer ses responsabilités et rejeter cette ordonnance. Tout le reste n'est que de la mascarade ! On gesticule pour faire croire que l'on fait quelque chose ici. Mais quel que soit le vote

est à Mme la ministre. Je continue d'affirmer que cette réforme est nécessaire. Elle a été promise par tous les gouvernements qui nous ont précédés.